amendement. Dans un souci de simplification, le Gouvernement a proposé que l'habilitation des officiers de police judiciaire, les OPJ, ne soit plus renouvelée à chaque fois qu'ils changent d'affectation. Le présent amendement tend à prévoir un renouvellement de l'habilitation tous les dix ans, afin de garantir, comme l'a indiqué Jacques Bigot, un contrôle régulier de l'autorité judiciaire. Cette proposition figurait dans le rapport Beaume-Natali. Cette formalité supplémentaire n'a pas paru nécessaire à la commission des lois pour garantir le contrôle de l'autorité judiciaire qui s'exerce surtout par le biais de la notation des OPJ par les procureurs généraux et du contrôle qu'exerce la chambre de l'instruction,

En pratique, la demande d'autorisation implique actuellement que l'officier de police judiciaire rende compte de l'avancée de l'enquête auprès du magistrat. Il est donc permis de s'interroger sur l'intérêt opérationnel d'une telle mesure. Par ailleurs, la présence d'un officier de police judiciaire territorialement compétent est aujourd'hui imposée par l'article 18 du code de procédure pénale lors des opérations réalisées par les enquêteurs hors de leur ressort, afin de permettre la prise en compte de toute situation imprévue. L'article 30 du projet de loi prévoit de rendre cette exigence facultative, à la discrétion du magistrat. Cette disposition risque de créer des situations procédurales et opérationnelles particulièrement dommageables, par exemple en cas de découverte incidente ou inopinée de stupéfiants ou d'armes au cours d'une perquisition. C'est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer les alinéas 5 et 6 de l'article 30. de la commission ? Le texte prévoit de faciliter le déplacement des OPJ sur le territoire national : au lieu d'imposer une commission rogatoire du juge d'instruction ou une réquisition du procureur, une simple information de ces magistrats suffira pour que l'OPJ poursuive son enquête en dehors des limites de son lieu d'exercice habituel. La commission des lois a estimé que cette évolution était positive. Comme c'est déjà le cas, le juge d'instruction ou le procureur pourrait exiger

en période estivale ou de pallier une absence d'effectifs. Sa finalité a depuis évolué et, sous l'autorité de leur commandant d'unité, les réservistes effectuent à présent des missions en autonomie dans le cadre d'un détachement de surveillance et d'intervention. Ils sont alors des entités opérationnelles à part entière et peuvent notamment être amenés, en tant que primo-arrivants, à constater des crimes, délits ou contraventions et à en dresser procès-verbal. Le problème vient du fait que cette compétence est exclue pour ceux d'entre eux qui sont recrutés au sein de la société civile. Ils sont légalement limités à la qualité d'agents de police judiciaire adjoints, en application de l'article 21 du code de procédure pénale, qualité judiciaire insuffisante au regard de l'évolution de leur emploi.

Au même grade, un sous-officier de réserve devrait en effet avoir accès à la même qualité judiciaire, et ce peu importe l'origine de son recrutement, à partir du moment où il répond aux exigences de connaissances requises pour accéder à la compétence De plus, la direction générale de la gendarmerie nationale a mis en place la formation de jeunes officiers de réserve, majoritairement issus de la société civile, appelés à commander aussi bien les personnels venant de la société civile que ceux qui ont fait leur carrière au sein de la gendarmerie nationale. Il paraît ainsi doublement contradictoire que ces officiers ces officiers de réserve soient, sur un plan militaire, leurs supérieurs et, sur un plan judiciaire, leurs subordonnés, alors que, pour les gendarmes de carrière, la qualité judiciaire conditionne la progression hiérarchique. C'est pourquoi, afin de gagner en logique, en clarté et en efficience, nous proposons cet amendement qui permet l'accès à la qualité d'APJ aux sous-officiers et officiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie. En concertation avec la direction générale de la gendarmerie nationale, il appartiendra au pouvoir exécutif, par décret en Conseil d'État, de fixer les conditions d'accès à cette qualité judiciaire, et donc à l'un de ces deux corps. Cela pourrait se faire par l'obtention d'une certification, à la suite d'un contrôle de connaissances. Leur apprentissage aurait alors lieu à distance avec pour obligation de préparer l'examen à partir de la plateforme en ligne GendForm 3.0, qui a été élaborée par la gendarmerie nationale depuis plusieurs années et qui a fait ses preuves. L'épreuve réussie, le réserviste pourrait alors accéder au corps des sous-officiers ou officiers de réserve, condition nécessaire pour devenir APJ. Quel est l'avis de

Aux termes des articles 20 et 20-1 du code de procédure pénale, sont déjà APJ les gendarmes servant dans la réserve.

procéder à des prélèvements, recourir à une personne qualifiée pour des examens techniques ou scientifiques, requérir des informations auprès d'organismes publics. Ensuite, ces actes sont effectués, dans le cadre de l'enquête préliminaire, sur autorisation du procureur de la République, ce qui constitue du point de vue de la commission

amendement tend à préciser que ces derniers agiront alors sous le contrôle des officiers de police judiciaire. Cet amendement ne me paraît pas justifié pour deux raisons lors de l'enquête préliminaire, l'OPJ ou l'APJ pourront, en principe, effectuer des réquisitions uniquement sur autorisation du procureur de la République

Ces dispositions constituent en effet une simplification de la procédure. En outre, elles ne remettent nullement en cause les garanties qui sont offertes dans ce domaine, en particulier le droit pour la personne gardée à vue de présenter des observations au procureur et l'obligation pour ce dernier de justifier de la nécessité de la prolongation de la garde à vue. Je rappelle que la présentation obligatoire, sauf à titre exceptionnel en cas de décision du magistrat de prolonger sans présentation préalable, n'existe que depuis la loi relativement récente du 14 avril 2011. 2011. Cette loi a été adoptée pour mettre notre droit en conformité avec des exigences constitutionnelles et conventionnelles. Dans la décision QPC du 30 juillet 2010 à l'origine de cette réforme, n'avait absolument pas critiqué le droit existant pour ce qui concerne les modalités d'intervention du procureur en matière de prolongation

à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet et que le déroulement de la garde à vue était placé sous le contrôle du procureur de la République pouvant décider, le cas échéant, de la prolongation de vingt-quatre heures. Le Conseil constitutionnel avait jugé que ces dispositions ne méconnaissaient en aucune manière l'article 66 de la Constitution. Voilà la raison pour laquelle je souhaite rétablir les dispositions relatives à la garde à vue telles qu'elles figuraient dans le projet de loi initial.

dans lesquels il sera procédé sur les lieux du transport à des actes pour lesquels la personne peut être assistée par un avocat, c'est-à-dire les cas d'audition, de reconstitution ou de tapissage. La commission des lois a ajouté l'hypothèse des transports pour procéder « à de nouvelles constatations ou saisies ». Cela ne me paraît pas justifié, car rien n'exige qu'un avocat soit présent lorsque les enquêteurs procèdent à des constatations ou à des saisies. Dans de tels cas, la personne suspecte est simplement présente, mais elle n'est pas interrogée.

Monsieur le corapporteur,

qui a contribué à accorder de nouveaux droits à la défense au stade de l'enquête. Depuis cette réforme, la victime peut être assistée de son avocat lors de la confrontation avec l'auteur de l'infraction. Si cela constitue un progrès, il est nécessaire d'aller plus loin et de lui permettre d'être assistée par un avocat dès le dépôt de plainte et pour toutes les auditions qui suivront. Cette réforme a même été une demande du principal syndicat de magistrats,

et lors des auditions peut être utile à une victime. Car les dépositions de celle-ci peuvent être maladroites ou inexactes du fait de l'émotion ou du traumatisme vécu ; l'assistance d'un avocat peut donc être indispensable pour éviter une erreur judiciaire dans laquelle la véritable victime ne sera pas reconnue comme telle. conséquent proposé de modifier le dispositif juridique de l'enquête de flagrance et de l'enquête préliminaire, d'une part, en informant obligatoirement la victime de son droit d'être assistée par un avocat dès le dépôt de plainte et lors de toute audition par les forces de l'ordre prévoyant les modalités concrètes de la présence de l'avocat auprès de la victime- droit de poser des questions à la fin de l'audition et de présenter des observations écrites versées au dossier. Les frais liés à l'assistance de l'avocat ne pourraient être pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle.

de son droit d'être assistée par un avocat dès le dépôt de sa plainte et lors de toute audition au cours de l'enquête. L'amendement vise également à préciser que l'avocat pourra poser des questions à la fin de l'audition de la victime et présenter des observations écrites versées au dossier. Il me semble que les modifications proposées sont satisfaites par le droit existant depuis la loi du 17 août 2015, qui a transposé la directive sur les droits des victimes

émettra un avis défavorable.

la poursuite des opérations policières et judiciaires dans une langue maîtrisée par l'individu, et non plus dans la langue qu'il déclare comprendre. J'avais déjà alerté le ministre de l'intérieur, le 20 juin dernier, lors de la discussion du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile En effet, actuellement, lors de l'interpellation d'un étranger déclarant comprendre uniquement une langue rare, il est légalement impossible d'accomplir les investigations, puisque les forces de l'ordre ne peuvent procéder ni à la notification des droits dans le cadre d'une garde à vue ou d'une audition libre ni à une audition dans la langue que la personne déclare comprendre. étranger comprendrait manifestement une autre langue, la procédure judiciaire doit se poursuivre dans la langue initialement déclarée par ce dernier. sur le fait que, en l'état actuel des textes, tant les forces de sécurité que les officiers de police judiciaire se heurtent à une carence importante en matière d'interprètes agréés, désignés d'ailleurs par des juridictions. Quel

effet, les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale résultent de la transposition, par la loi du 27 mai 2014, des exigences de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales. De ce fait, il n'est pas possible, à cadre européen constant, de faire droit

En effet, contrairement à ce qui figure dans l'objet de l'amendement, la notification des droits peut déjà avoir lieu dans toute langue maîtrisée par la personne, et non seulement dans la langue qu'elle déclare comprendre. D'autre part, la notion de langue officielle de son pays d'origine ou de toute autre langue officielle ne correspond pas forcément à une langue que la personne comprend. Aussi, passer

une autre étape permet de définir une langue qu'elle peut effectivement maîtriser. Il est inutile de vous dire que, dans le contexte des phénomènes de migration que nous pouvons connaître sur le territoire de Calais,

à la mise en place de plateformes de traduction pour les langues peu usitées, ce qui, nous l'espérons, nous permettra d'avoir plus de souplesse sur ces questions.

Il octroie aux policiers, sans garde-fous, des pouvoirs d'écoute, de géolocalisation et de perquisition pour une multitude de délits qui n'ont rien à voir avec le grand banditisme ni avec le terrorisme. Il fait ainsi entrer encore davantage l'état d'urgence dans l'état de droit. La justice repose sur le principe de la balance entre l'accusation et la défense ; sans cet équilibre, vous n'avez plus de justice. C'est ainsi la conception même de la justice qui est menacée. L'article 32 étend les pouvoirs des enquêteurs au travers de l'intégration dans le droit commun des dispositifs actuellement prévus pour la seule poursuite des délits donnant lieu à une peine de prison de plus de cinq ans ou des infractions de terrorisme ou de criminalité organisée. Les pouvoirs exceptionnels confiés aux enquêteurs dans le cadre de l'enquête de flagrance, qui sont justifiés par un crime ou par un délit qui vient d'être commis, n'ont aucune raison d'être étendus à un autre cadre juridique. En effet, ces pouvoirs ne sont justifiés que par « la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité », conformément à l'article 54 du code de procédure pénale. nécessaire de réfléchir à la restriction de ce régime dérogatoire de l'enquête de flagrance à une durée strictement limitée à l'urgence, le projet de loi prévoit au contraire son extension et sa banalisation par deux moyens. l'extension de la durée de la flagrance à seize jours lorsque la procédure porte sur un crime de droit commun ou sur une infraction prévue, entre autres, par l'article 706-73 part, de l'extension de la possibilité de prolonger la flagrance à l'ensemble des infractions punies de trois ans d'emprisonnement ou plus. Or la formulation de cette disposition et la confusion de l'étude d'impact ne permettent pas d'exclure tout à fait formellement une application aux crimes de droit commun et aux infractions prévues par l'article que je viens de citer. Pour toutes ces raisons, nous souhaitons la suppression du présent article particulièrement attentatoire aux libertés fondamentales, alors que, en parallèle, une réduction sensible de l'autorité judiciaire est à l'oeuvre. La parole

précédents : les pouvoirs exceptionnels confiés aux enquêteurs dans le cadre de l'enquête de flagrance, justifiés par la nécessité de la « conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à manifestation de la vérité », sont ici largement élargis. Il peut s'agir d'une perquisition sans l'assentiment de la personne, d'une perquisition de nuit ou d'une interdiction d'éloignement. Toutes ces mesures obéissent au critère de l'urgence, qui, par définition, n'existe que dans une période limitée. Seule la limitation stricte de cette période permet que les atteintes à la liberté individuelle soient encadrées par les principes de nécessité et de proportionnalité issus de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

En effet, afin d'améliorer l'efficacité des enquêtes, les dispositions de l'article 32 adaptent la durée de l'enquête de flagrance à la réalité et aux besoins du terrain, et elles abaissent le seuil des perquisitions autorisées par le juge des libertés et de la détention dans le cadre Ces modifications que je propose nous semblent justifiées. Ainsi, la fixation d'un seuil de trois ans au lieu de cinq permettant de prolonger l'enquête de flagrance de huit jours ou pour autoriser la réalisation d'une perquisition sans l'assentiment de la personne concernée atteste d'une certaine gravité de l'infraction. Je le rappelle, les délits punis de trois ans d'emprisonnement sont les délits de soustraction d'un mineur par un parent, de vol- je pense par exemple

ces durées représente un intérêt opérationnel indéniable, notamment pour les faits de soustraction d'un mineur par ascendant, dont je viens de parler, ou bien d'abus de confiance, qui peuvent porter sur des préjudices extrêmement importants. De même, le fait de porter la durée de l'enquête de flagrance de huit à seize jours en matière de criminalité et de délinquance organisées, sans qu'il soit nécessaire, comme c'est actuellement le cas, d'en faire ordonner la prolongation par le procureur de la République, se justifie par l'urgence qu'il y a à poursuivre des actes d'investigation et à disposer et à disposer de pouvoirs de contrainte pour ces faits d'une particulière gravité. Il nous semble, enfin, que les modifications que nous proposons ne portent pas une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales, parce que la perquisition est autorisée par le juge des libertés et de la détention- je ne reviens pas sur ce que nous avons dit tout à l'heure à ce Par ailleurs- cela entre toujours dans l'équilibre des droits -, le projet de loi renforce le contrôle opéré par le procureur en obligeant celui-ci à rendre une décision écrite et motivée pour prolonger la flagrance. D'autre part, ceci est tout à fait nouveau- c'était demandé par le Conseil d'État -, le texte reconnaît désormais aux personnes non poursuivies le droit de contester la légalité, la régularité d'une perquisition devant le JLD, six mois après la perquisition. Selon moi, l'ensemble des garanties ainsi énoncées équilibre le texte.

l'extension, non négligeable, des durées prolongées de l'enquête de flagrance, dès lors qu'elle semble de moins en moins caractérisée par l'urgence, de moins en moins placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire et susceptible de concerner la quasi-totalité des délits, même mineurs ». Vous rappelez ensuite que « la jurisprudence constitutionnelle déduit de l'article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire et que celle-ci doit assurer le contrôle " direct et effectif " des officiers de police judiciaire.

La loi du 9 mars 2004 a prévu la possibilité d'une prolongation de l'enquête par le procureur de la République- huit jours supplémentaires -pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement.

1 à 4, au nom du respect de nos règles de droit et de la Constitution.

Ces dispositions constituent en effet une complexification majeure de la procédure pénale, qui n'est pas, en tout cas à ce jour, imposée par les exigences européennes.

et opérations de reconstitution et de tapissage. En outre, on voit assez mal la manière dont pourraient s'appliquer en pratique Il faudrait peut-être attendre pendant deux heures un avocat avant de commencer la perquisition, comme cela est prévu pour l'assistance de l'avocat pendant l'audition du gardé à vue. Cette attente devrait-elle se répéter à chaque perquisition sur des lieux différents, si plusieurs perquisitions sont réalisées à la suite, dans la même journée,

Aurait-il fallu attendre l'appel de l'avocat puis sa venue pour pouvoir réaliser cette perquisition ? Je n'en suis pas sûre. Quel serait, enfin, le rôle de l'avocat lors de cette perquisition ? Par définition, au moment de la perquisition, la personne n'est pas interrogée. La régularité de la perquisition est attestée par des procès-verbaux que la personne présente est invitée à signer et non par la présence de l'avocat. Il me semble donc que ce processus n'est pas compatible avec les exigences des enquêtes, et c'est d'ailleurs bien la raison pour laquelle la directive européenne précitée, pourtant très

lors que, petit à petit, la place du juge d'instruction est moins importante et que celle du procureur diligentant les enquêtes le devient de plus en plus, il est indispensable de recréer le respect du contradictoire

de M. Grosdidier sur l'état des forces de sécurité intérieure. Cette commission relevait largement le découragement des enquêteurs devant les lourdeurs procédurales.

contribuerait à créer encore une tâche supplémentaire pour les enquêteurs. C'est exactement l'opposé de ce que je vise. La

la grande majorité des amendements que vous présentez, permettez-moi de vous le dire en toute simplicité, visent à revenir au texte initial du projet de loi. Ce caractère quelque peu systématique finit par poser

d'amendements tendant à revenir au texte initial, qui serait souverainement bon, a quelque chose d'un peu caricatural, et, je le sais, madame le garde des sceaux, vous n'aimez pas du tout ce qui est caricatural, je vous donne acte

est à M. Jacques Bigot. Chers collègues rapporteurs, vous êtes bien récompensés par Mme la garde des sceaux d'avoir fait des efforts pour essayer de sauver cet article 32,

pense et écrit la commission des lois. Sans doute en raison de quelque inadvertance n'avez-vous pas observé que j'ai déjà pris en compte un certain nombre de remarques. Je pense notamment à l'obligation de motivation écrite dont

matière pénale : lorsque la peine encourue est d'au moins trois ans, par exemple, le magistrat n'a pas à contrôler la double incrimination pour exécuter un mandat d'arrêt européen ; de même, il ne peut refuser d'exécuter

Mme la garde des sceaux. Cet amendement tend à rétablir la possibilité pour les enquêteurs de pénétrer au domicile d'un suspect afin de l'interpeller dans le cadre d'un ordre à comparaître délivré par le parquet. Cette possibilité a été supprimée par la commission des lois au motif que les enquêteurs peuvent pénétrer au domicile d'un suspect dans le cadre d'un mandat de recherche délivré par le parquet. Ce raisonnement, même si je peux l'entendre, ne me semble pas satisfaisant. Je rappelle que la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, adoptée par le Sénat, a permis au procureur d'autoriser les enquêteurs à faire comparaître un témoin ou un suspect par la force publique.

Le projet de loi vient donc combler cette lacune en permettant une telle introduction au domicile des suspects lorsque la peine encourue est d'au moins trois ans. En refusant cette simplification, votre commission complique inutilement la tâche des magistrats et des enquêteurs. En effet, dans un tel cas, soit les parquets délivreront systématiquement des mandats de recherche, même lorsque le domicile du suspect est connu- ce qui, avouons-le, est quelque peu curieux

Il me semble qu'il serait plus sage que le Sénat, dans la continuité des textes adoptés en 1993 et en 2004, accepte cette simplification de bon sens. Très belle argumentation

Dans le cadre de contrôles et de vérifications, certains agents de police judiciaire adjoints, ou APJA, sont déjà autorisés à assister les officiers de police judiciaire pour diverses opérations- contrôle d'identité, visite de véhicule ou fouille de bagages. Il s'agit des adjoints de sécurité, ou ADS, de la police nationale et des gendarmes adjoints volontaires, ou GAV. Afin d'optimiser la qualité des services rendus par les policiers municipaux, nous proposons d'autoriser également ces derniers à effectuer ces différents contrôles sous l'autorité d'un OPJ

Alors que l'objectif affiché des dispositions de l'article 32 est la simplification des régimes, nous nous sommes interrogés sur la pertinence de créer un nouveau régime permettant de forcer un domicile dès lors que l'article 77-4 du code de procédure pénale prévoit déjà la possibilité de pénétrer pendant la même plage horaire dans un domicile pour exécuter un mandat de recherche délivré par le procureur de la République « contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre » un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement. L'étude d'impact souligne d'ailleurs que les conditions de recours à cette procédure sont identiques à celles du mandat de recherche : une peine encourue d'au moins trois ans d'emprisonnement et une décision préalable d'autorisation par le procureur de la République écrite et motivée. La création de ce régime nouveau s'ajoute donc au panel des possibilités, alors que la délivrance d'un mandat de recherche est déjà possible, même lorsque le domicile de la personne convoquée est connu.

que la participation des agents municipaux à un dispositif administratif de prévention des troubles à l'ordre public obligeait à ce que les officiers de police judiciaire assurent un contrôle effectif et continu sur ces personnes, ce qui exclut toute action autonome de leur part et donc limite la portée d'une telle disposition. Ces propos prennent un sens tout particulier dans la période que nous traversons. En l'état de l'organisation de l'autorité judiciaire, de la formation inégale des policiers municipaux et des articulations disparates entre les dispositifs de la police nationale et de la police municipale, il paraît prématuré de proposer que des policiers municipaux puissent effectuer des contrôles d'identité. Par ailleurs, les dispositions des articles 78-2-3 et 78-2-4 du code de procédure pénale donnent des pouvoirs autonomes à l'officier de police judiciaire qui agit d'initiative, et non pas en exécution de réquisitions du procureur de la République. Il ne semble pas possible de confier à des policiers municipaux un pouvoir d'initiative en matière de contrôles d'identité ou de fouille de bagages. Je tenais à être précis sur ce sujet extrêmement important.

pas précisé que cette procédure quelque peu particulière s'appliquait non seulement au domicile de la personne qu'il convient de faire comparaître, mais également à tous les lieux où elle est susceptible de se trouver. En clair,

Alors que cette présence est prévue dans le code de procédure pénale pour les visites domiciliaires, un vide juridique subsiste quant à la possibilité pour celui-ci d'être présent lors de la perquisition pénale. Nous proposons ainsi de mettre fin à cette absence et aux incertitudes qui en résultent, notamment au regard de la législation européenne. En effet, la directive 2013/48 de l'Union européenne relative aux droits du justiciable énonce qu'avant qu'ils soient interrogés par la police, ou par une autre autorité répressive ou judiciaire, les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat sans retard indu. Au-delà de la mise en conformité avec le droit communautaire, la présence de l'avocat, auxiliaire de justice, est une mesure de bon sens contribuant à la transparence et au bon déroulement de la perquisition- elle ne saurait, de ce fait, être perçue comme une obstruction à la procédure pénale et judiciaire -et permettant de prévenir

de plus en plus de Français s'approvisionnent à l'étranger ou sur le marché parallèle au détriment des buralistes, très fortement affectés. L'Office européen de lutte antifraude, ou OLAF, précise que la contrebande de tabac entraîne chaque année des pertes importantes pour les budgets des États membres et de l'Union européenne, sous la forme de droits de douane et de taxes éludés. Les ventes de tabac de contrebande ne respectent aucune règle et représentent un risque considérable pour les consommateurs et les entreprises. Elles nuisent aux campagnes de santé publique et de lutte contre le tabagisme et enfreignent les règles strictes que l'Union européenne et les États membres ont fixées concernant la fabrication, la distribution et la vente. Ainsi, la contrebande de cigarettes et des autres produits du tabac est un phénomène mondial qui, au sein de l'Union européenne seule, entraîne une perte annuelle de plus de 10 milliards d'euros de recettes fiscales. Très rentable, facile à mettre en oeuvre et peu risqué, le commerce illicite de tabac de contrebande s'accroît. Il constitue un terreau propice à la marginalisation sociale et à la délinquance, mais surtout alimente considérablement le terrorisme et le crime organisé. Selon le rapport du 30 mars 2015 du Centre d'analyse du terrorisme, « la contrebande et le trafic de cigarettes représentent plus de 20 % des sources criminelles de financement des organisations terroristes », un phénomène qui prend de l'ampleur depuis l'an 2000.

Certaines des pistes de réforme de la procédure pénale, remontées par les agents des forces de sécurité intérieure, paraissent mériter une attention particulière.

à faire de certains enregistrements audio des pièces de procédure à part entière qui seraient versées au dossier, au même titre qu'une pièce écrite, éventuellement accompagnées d'un procès-verbal de synthèse. Rien ne permet en effet de postuler que seule la forme écrite écrite garantit le formalisme de la procédure, dont le respect peut être aussi garanti par un enregistrement sécurisé. Si une oralisation totale des procédures paraît exclue à ce stade, l'oralisation de certains actes de procédure, dans le cadre de procédures simples,

exprimée lors des auditions menées par la commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité. Voilà, madame le garde des sceaux, une proposition concrète d'allégement du fardeau procédural des forces de sécurité. Quel

il ressort de toutes les consultations que j'ai pu conduire que cette oralisation ne fait pas du tout l'unanimité au sein des services de la police et de la gendarmerie. Elle est aussi vivement critiquée par les magistrats et les avocats. En effet, si le fait de procéder à un enregistrement audio accompagné d'une synthèse écrite, au lieu de rédiger un procès-verbal complet,

pour réellement mettre en place des procédures simplifiées. Je pense, par exemple, au procès-verbal unique, qui existe déjà, mais qui n'est pas toujours utilisé par les services enquêteurs. Nous avons donc décidé, avec le directeur des affaires criminelles et des grâces avec les services du ministère de l'intérieur, de créer des fiches pratiques que nous allons diffuser à l'ensemble des enquêteurs et qui, je l'espère, nous permettront de mettre en place des méthodes de travail simplifiées.

Cet amendement vise à pouvoir considérer juridiquement les données issues d'objets connectés dans le cadre d'une enquête judiciaire, au titre de l'accusation ou de la défense.

De nombreux objets connectés permettent en effet de connaître la géolocalisation, le rythme cardiaque, ou encore l'utilisation des appareils électroniques d'un lieu donné. Il est donc nécessaire que ces éléments matériels puissent être mobilisés devant une cour, dans le cadre d'une accusation ou d'une défense. En droit français, le principe est que la preuve admissible est libre en matière civile- à l'exception d'actes tels que des contrats -, administrative et pénale, ce qui offre aux avocats ou aux procureurs la possibilité de produire de telles données devant un tribunal à l'appui de leurs demandes. Ils peuvent aussi solliciter du juge une ordonnance judiciaire pour obtenir des prestataires les données collectées concernant la partie adverse ou un tiers au procès, si de telles données peuvent éclairer le tribunal. Dans le cadre des enquêtes policières, la loi précitée prévoit déjà la possibilité pour la police judiciaire d'utiliser « tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel ce qui avait été clairement établi lors des débats, comme la possibilité de géolocaliser n'importe quel objet connecté, soit directement par ses coordonnées GPS, s'il en émet, soit par le truchement des réseaux fixes ou mobiles auxquels il est connecté.

en effet d'introduire un élément de rigidité, là où il convient de préserver une certaine souplesse dans l'appréciation au cas par cas des relations qui peuvent exister entre la personne mise en cause et les magistrats susceptibles de juger l'affaire ou les fonctionnaires de la cour d'appel.

En tant qu'agents de police judiciaire adjoints, ou APJA, les policiers municipaux ne peuvent aujourd'hui que constater l'existence d'un état alcoolique, sous la responsabilité d'un OPJ, sans pouvoir procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique par la mesure précise de la concentration d'alcool dans le sang. En cas de présomption de l'existence d'un état alcoolique, ils doivent en rendre compte immédiatement à tout OPJ territorialement compétent, qui peut ordonner la présentation sur-le-champ de la personne concernée. Ils doivent ainsi transporter l'individu auprès d'un OPJ. En pratique, ils se voient confier par l'OPJ les vérifications du taux d'alcoolémie. Ainsi, ils peuvent donc être mobilisés plusieurs heures pour la procédure.

Entre 0,5 gramme et 0,8 gramme, les APJA pourraient directement établir l'amende. Il s'agit là d'une véritable simplification permettant de mieux lutter contre l'alcool au volant.

Concernant les règles relatives aux contrôles d'alcoolémie et d'usage de stupéfiants sur les conducteurs, il prévoit de confier aux agents de police judiciaire, les APJ, la possibilité de prendre seuls l'initiative d'un contrôle. En l'état du droit, l'initiative des contrôles d'alcoolémie ou d'usage de stupéfiants sur les conducteurs est prise soit sur instructions du procureur de la République, soit sur l'initiative d'un officier de police judiciaire. Le contrôle peut alors être effectué alors être effectué par des APJ ou des agents de police judiciaire adjoints, sur les instructions et sous la responsabilité de l'officier de police judiciaire. La mesure proposée par l'article 33 du projet de loi n'est pas neutre. Elle permettrait notamment à un élève gendarme ou à un policier stagiaire de prendre seul, sans supervision ni contrôle d'un professionnel de plein exercice, l'initiative de contrôles routiers d'alcoolémie. Le fait de confier l'initiative de ces contrôles aux APJ, qui justifient d'un niveau de formation procédurale moindre et font l'objet d'un contrôle plus réduit, risque de fragiliser la qualité procédurale des opérations menées. Nous estimons donc qu'il convient d'en rester au au niveau de garantie assuré par le droit en vigueur, les agents de police judiciaire pouvant d'ores et déjà être chargés de la réalisation concrète des opérations. Seuls l'initiative et le contrôle d'un officier de police judiciaire sont requis par la loi. Quel

extrêmement attendue par l'ensemble des acteurs de terrain. Elle a même fait l'unanimité lors de la consultation des praticiens dans le cadre des chantiers de la justice, comme l'ont d'ailleurs relevé MM. Beaume et Natali, qui ont rédigé le rapport auquel il a été fait plusieurs fois allusion.

allant parfois jusqu'à dénaturer les textes applicables. La position qui prédomine repose sur une appréciation purement générale et abstraite des critères de la légitime défense. Or elle paraît totalement déconnectée des situations de violence et des réalités du terrain. Plusieurs droits étrangers privilégient au contraire une conception plus pragmatique et réaliste du droit de la légitime défense, en considérant l'état dans lequel se trouvait la victime quand elle a riposté. En Allemagne, la notion de peur est prise en compte. L'article 33 du code pénal allemand énonce que « si par désarroi, crainte ou terreur, l'auteur dépasse les limites de la légitime défense, il n'est pas puni En Suisse, l'article 16 du code pénal helvétique prévoit que la victime n'a pas agi de manière coupable, si, en repoussant une attaque, elle a excédé les limites de la légitime défense dans « un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque Cet amendement vise à adapter le droit de la légitime défense aux contingences de la réalité contemporaine, notamment à celles que connaissent les commerçants agressés sur leur lieu de travail. L'explosion de la délinquance violente et la multiplication des actes de défense excusables imposent de faire évoluer notre droit et de prendre en compte, parmi les critères d'évaluation de la légitimité des actes de défense, l'état de la victime causé par la nécessité de se défendre en situation vitale. Le présent amendement vise donc à insérer à l'article 122-5 du code pénal, parmi les critères d'évaluation de la légitimité des actes de défense, la prise en compte de l'état de la victime au moment de sa riposte. Modernisons-nous un peu ! Quel est

explication de vote. Naturellement, nous sommes obligés de respecter la motivation de nos collègues qui ont déposé cet amendement, parce que le sujet est réel. Le policier, la personne des forces de l'ordre placée dans une situation d'agression et de réplique immédiate, peut commettre

pour faire face à une agression dans son commerce ? Est-il légitime de tuer soi-même un délinquant, alors qu'il n'y a pas de proportionnalité entre la réplique

sur la nécessité de ne pas donner aux procureurs de pouvoirs excessifs. Nous devons en effet respecter un certain nombre de principes fondamentaux de notre République. Je crains fort

votre présentation, en indiquant qu'il existe déjà dans notre législation toute une série de dispositifs permettant de prendre en compte les états que vous évoquez.

Les présomptions de légitime défense sont souvent dévoyées par la jurisprudence. Or une telle position paraît totalement déconnectée des situations de violence et des réalités du terrain. Cet amendement vise à adapter le droit de la légitime défense aux contingences de la réalité contemporaine, notamment

envisage la création d'un tribunal criminel, afin de désengorger notamment de ce type de contentieux les cours d'assises. L'explosion de la délinquance violente et la multiplication des actes de défense excusables imposent de faire évoluer notre droit et d'élargir ainsi les cas de présomption de légitime défense. Il convient tout d'abord de sanctuariser le domicile. Là où la loi n'offre une présomption de légitime défense que « pour

a légitime défense lorsque quelqu'un vient porter atteinte à votre intégrité physique et que vous réagissez

La nuit, vous ne saviez pas que la personne n'avait pas de couteau ou de pistolet et vous avez tiré : vous êtes dans un cas de présomption de légitime défense.

ou la cour d'assises que vous étiez bien en situation de légitime défense. Je crois que c'est assez normal, que notre loi n'est pas si mal faite et que le Parlement, qui a déjà eu l'occasion de délibérer de ces questions à de nombreuses reprises, ne fait pas toujours si mal son travail. Nous ne sommes pas aussi démunis qu'on pour faire face aux difficultés. C'est la raison pour laquelle je suis d'accord pour rechercher le plus possible de nouvelles règles qui nous permettent de mieux lutter contre la délinquance

que vous ne voudriez pas voir opposer à votre fils, à votre frère ou à votre neveu. Prenons garde à ce que les règles restent bien équilibrées, même si la ligne directrice de notre politique est quand même

corapporteur. Je veux dire à M. Reichardt, qui m'a interpellé tout à l'heure, qu'à mon tour je l'incite

Monsieur Duplomb, la jurisprudence et le texte que vous avez évoqués tout à l'heure pour les agressions et les intrusions de nuit sont constants

La période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal repose sur l'idée que la cour d'assises, au vu de la gravité des faits, de la personnalité de l'accusé et des risques de récidive, doit pouvoir s'assurer qu'une partie au moins de la peine d'enfermement qu'elle prononce sera exécutée avec certitude, sans aucune libération anticipée possible. Dès lors qu'une marge d'appréciation de la juridiction d'application reste possible pour le restant de la peine prononcée, rien ne justifie que celle-ci puisse également écarter ou réduire la période de sûreté.

Dans sa décision du 20 janvier 1994, le Conseil constitutionnel a rappelé que l'exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion. le Conseil n'a pas déclaré la peine de perpétuité incompressible, prévue par les dispositions des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, contraire au principe de nécessité des peines, c'est en raison de la procédure prévue justement par les dispositions de l'article 720-4 du code de procédure pénale, qui permet le réexamen de la situation du condamné par le tribunal de l'application des peines à titre exceptionnel et à l'issue d'une période minimale de trente ans, lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale. De plus, si l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme n'interdit pas aux États d'infliger des peines perpétuelles aux auteurs d'infractions graves, la Cour européenne, quant à elle, exige que soient prévues la possibilité d'un réexamen et une chance d'élargissement de la peine au moins après trente L'impossibilité d'un réexamen par l'autorité judiciaire de la peine dans la perspective de la commuer, de la suspendre, d'y mettre fin ou de la poursuivre, est contraire aux dispositions de l'article 3

Nous faisons en effet le constat d'un droit résiduel en matière d'information de l'avocat pendant la garde à vue. Or, d'une manière générale, l'équité d'une procédure pénale requiert que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment où il est placé en garde à vue. Ainsi, il s'agit d'améliorer l'accès au dossier dès le début de la procédure, tant pour le prévenu que pour l'avocat. Cet amendement vise tout d'abord à renforcer les droits de la

ou des observations avant toute décision définitive du ministère public. De manière concrète, le procureur de la République devra aviser les parties de la mise à disposition d'une copie de la procédure et de la faculté de formuler des observations. observations. Le présent amendement tend également à permettre à l'avocat de disposer de l'accès au dossier de la procédure dès la garde à vue de son client. Il faut le rappeler, le droit d'accès de l'avocat aux pièces du dossier est prévu par l'article 7 de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012, dès lors qu'une personne est arrêtée et détenue à n'importe quel stade de la procédure pénale.

naturellement attachés aux droits de la défense, ainsi que nous l'avons démontré à l'occasion de l'examen de ce texte. Il faut cependant être attentif à concilier cette préoccupation avec celle de l'efficacité et de la rapidité des enquêtes, en veillant à ne pas dupliquer au stade de l'enquête préliminaire le formalisme prévu dans le cadre des informations judiciaires.

constitue, de mon point de vue, une complication importante de la procédure pénale qui, je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas exigée par les textes européens et, plus particulièrement, par la directive déjà citée du 22 mai la directive déjà citée du 22 mai 2012. Par ailleurs, la modification introduite par votre amendement, madame la sénatrice, conduit à une différence assez peu justifiée entre la personne qui est assistée d'un avocat et qui, dès lors, aurait accès à son entier dossier, et celle qui, n'étant pas représentée, n'aurait accès qu'à certaines pièces de la procédure. En outre, la systématisation du contradictoire à la clôture de l'enquête ajoute une forme de rigidité et de lourdeur qui s'inscrit à rebours de l'objectif de simplification et d'efficacité Alors que dans le souci d'une bonne administration de la justice, le projet de loi que je défends favorise une clôture de l'instruction plus rapide, votre amendement tend au contraire à imposer systématiquement au parquet d'attendre un mois avant d'engager des poursuites lors de toute enquête, et ce alors même que les parties ne souhaiteraient faire aucune observation ou demande d'actes. Cette lourdeur est d'autant plus inutile, me semble-t-il, que la loi, plus particulièrement l'article 388-5 du code de procédure pénale, permet déjà aux parties de demander tout acte qu'elles estimeraient utile à la manifestation de la vérité après l'engagement des poursuites jusqu'à l'audience. Je mets aux voix l'amendement

des lois, de poursuivre certains actes d'enquête, tels que les interceptions, les géolocalisations, les techniques spéciales d'enquête en cas d'ouverture d'une information pour toute infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement. Un tel « sas » ne doit pas être limité à la seule délinquance et criminalité organisée, comme le souhaite la commission des lois. En effet, ce sas, cette période, se justifie, non pas en raison de la nature de l'infraction, mais, au contraire, au regard de la nécessité d'éviter une discontinuité dans le déroulement des investigations. des investigations. En cas d'ouverture d'une information, ce sas permet ainsi d'assurer la poursuite sans interruption de l'interception téléphonique, de la géolocalisation, de la sonorisation ou de toute autre technique spéciale d'enquête.

Au bout d'un mois d'enquête infructueuse, il serait décidé d'ouvrir une information judiciaire : faut-il permettre que l'écoute lancée au moment de l'enquête cesse le temps que l'information soit ouverte avant que cette même écoute soit de nouveau ordonnée par le juge d'instruction ? Il y a là une discontinuité qui ne nous paraît pas utile et qui semble préjudiciable aux informations recueillies. Le mécanisme que je vous propose ne porte en rien atteinte aux prérogatives du juge d'instruction, puisque celui-ci pourra à tout moment décider de mettre fin aux mesures en cours. Il me semble donc que le sas est particulièrement utile et doit être rétabli.

Je rappelle que le Gouvernement considère qu'une telle disposition, qui permet de prolonger des techniques spéciales d'enquête ou des interceptions sans contrôle du juge du siège, est une mesure de simplification du travail du juge d'instruction, qui ne sera pas obligé de prononcer ces mesures en urgence. Néanmoins, si ces mesures sont urgentes et nécessaires, il semble tout de même logique que le magistrat chargé de l'enquête, à savoir le juge instruction, les prononce.

au moment même où il est saisi, peut décider d'arrêter ces mécanismes d'interception ou d'écoute. Il s'agit là d'une mesure de bon sens qui permet d'éviter la discontinuité, la rupture entre deux périodes juridiquement distinctes. Je trouve dommage de s'en priver. La parole est à M. le corapporteur. Je veux juste préciser à la Haute Assemblée que, en matière de terrorisme, cette possibilité est prévue pour une durée de

est non seulement superflu, mais constitue aussi une mesure déshumanisante et incompréhensible pour la victime qui se voit limitée dans l'accès au juge pénal. Aujourd'hui, en toute hypothèse, il est possible de déposer plainte avec constitution de partie civile, même sans avoir exercé de recours hiérarchique auprès du procureur général, contre la décision de classement sans suite prise par le procureur de la République. En outre, le juge d'instruction est tenu d'instruire une plainte avec constitution de partie civile, alors même que la totalité des investigations utiles à la manifestation de la vérité a déjà été réalisée par le parquet et que la partie civile aurait pu directement citer le prévenu devant un tribunal correctionnel. Or l'article 34 du projet de loi durcit considérablement les conditions d'exercice de la plainte avec constitution de partie civile dans les dossiers correctionnels en portant de trois à six mois le délai permettant au procureur de la République de répondre à une plainte simple avant que la victime ne puisse saisir le juge, et en ouvrant la possibilité au juge d'instruction de refuser l'ouverture d'une information judiciaire, lorsque celle-ci est inutile et qu'une citation directe de la victime est possible.

Il ne paraît pas déraisonnable de vouloir lutter contre les abus en matière de constitution de partie civile lorsque celle-ci paraît disproportionnée par rapport à l'intérêt public qu'elle représente, mais le droit en vigueur prévoit déjà des conditions strictes, directement inspirées par la volonté de réduire la charge occasionnée par certaines plaintes peu sérieuses. Une telle mesure est sans fondement et doit être rejetée.

Sincèrement, nous ne pouvons pas nier qu'il y a eu des abus en matière de constitution de partie civile. Il faut rappeler que les deux tiers des instructions ouvertes sur constitution de partie civile et clôturées en 2016 l'ont été par un non-lieu. Ce n'est Ce n'est quand même pas négligeable. L'allongement de trois à six mois du délai, qui permettra au procureur de la République de répondre à une plainte simple avant que la victime ne puisse saisir le juge, ne semble pas excessif à la commission des lois. De même, l'ordonnance de non-lieu informer nous paraît utile en cas de mesures alternatives aux poursuites qui ne conviennent pas aux victimes. Enfin, je rappelle que le texte de la commission a supprimé le recours préalable devant le procureur général. Quel est l'avis du Gouvernement ? Même avis

en principe, une juridiction ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Mais, par une construction jurisprudentielle, la Cour de cassation a établi de très nombreuses présomptions de grief. Elle considère ainsi que tout manquement à la règle de droit est, en lui-même, une cause de nullité de la procédure. Cette jurisprudence mérite à mon sens d'être infléchie en ce qu'elle va à l'encontre de l'esprit de la loi, qu'elle contredit l'objectif d'efficacité des procédures et qu'elle heurte le bon sens, avec parfois des remises en liberté de détenus totalement incompréhensibles. Quel

Je rappelle que, aux termes des dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale, il y a nullité seulement lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Ce point est important. L'obligation d'une démonstration systématique de toutes les nullités, même les plus évidentes, qui devrait en principe être relevée de plein droit par les juridictions de jugement, entraînerait des débats évidemment extrêmement fastidieux et un affaiblissement des garanties du justiciable. Imagine-t-on devoir démontrer la nullité d'une interception non autorisée par un juge ? Imagine-t-on devoir démontrer la nullité d'une autorisation de perquisition signée sept jours après la perquisition ? Naturellement, la réponse est non. C'est la raison pour laquelle la commission des lois émet un avis défavorable sur l'amendement n° 71 rectifié. Quel est

porté aux intérêts des parties et exigé en matière de nullité doit toujours être démontré et qu'il ne peut être présumé. L'objet de cet amendement est de contrecarrer la jurisprudence de la Cour de cassation, qui aurait établi de très nombreuses présomptions de grief. En réalité, il ne semble pas que cette modification changera l'état du droit, dès lors que la Cour de cassation ne pose pas de présomption de grief, mais constate que la violation de certaines formalités porte atteinte aux droits de la défense. De plus, si le Gouvernement entend effectivement simplifier la procédure pénale pour supprimer des formalismes inutiles, susceptibles d'entraîner actuellement des nullités, il ne souhaite pas envoyer comme message aux praticiens, notamment aux enquêteurs, que le non-respect des règles de procédure n'aurait plus de conséquences sur la régularité de celle-ci. Ce serait en effet une forme d'incitation à ne plus respecter la loi et nous ne voulons pas aller dans ce sens-là. C'est pourquoi j'émets un avis défavorable sur cet amendement.